La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2020 est parvenue à l'adoption d'un texte commun. la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (projet n° 114, texte

activité économique et financière : conformité des produits, gestion du Fonds européen agricole pour le développement rural, le Feader, protection des consommateurs, lutte contre le blanchiment d'argent. Il participe aussi au soutien de la culture, avec les dispositions relatives à la transposition des directives SMA- Services de médias audiovisuels - et Droit d'auteur. Cette diversité témoigne de l'importante activité normative des différentes instances de l'Union européenne, conduisant les États membres à adapter leur droit économique et financier à l'horizon des années 2020-2021. Ces adaptations auront un impact considérable. Je prendrai, à ce titre, deux exemples parmi d'autres. Tout d'abord, le projet de loi élargit le champ d'action des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Cette mesure est une avancée supplémentaire dans la protection de nos consommateurs.

à assujettir les plateformes installées à l'étranger aux obligations de financement de la production audiovisuelle et cinématographique, et, d'autre part, à garantir aux artistes une rémunération proportionnelle aux fruits de l'exploitation des oeuvres. La transposition de ces directives revêt aujourd'hui un caractère primordial pour les créateurs, dont les rémunérations ont été fortement affectées par la crise sanitaire. Ce projet de loi permettra également à notre pays, qui présidera le Conseil de l'Union européenne en 2022, d'être exemplaire en matière d'application du droit communautaire.

comme vous le savez, il subsiste un petit point d'achoppement dans les discussions que vous avez avec le Gouvernement. Le projet de loi comporte ainsi des dispositions issues de vos travaux. Je pense en particulier aux trois nouveaux articles concernant les vétérinaires, dont le dispositif de lutte contre la désertification vétérinaire, sur le modèle de la lutte contre les déserts médicaux.

Il est évidemment dommage que la commission mixte paritaire n'ait pu aboutir, en dépit d'un large consensus sur la plupart des mesures, faute d'accord sur le seul article 4 - j'imagine que nous y reviendrons -, qui reprenait la proposition de loi de la présidente Primas visant à garantir le libre choix du consommateur dans le cyberespace.

pensons notamment que celles-ci desserviraient la négociation européenne en cours. Ce projet de loi complexe comporte des dispositions multiples. Son objet est simple : faire évoluer la réglementation européenne, en la traduisant dans notre droit national. Ces avancées renforceront la protection de nos concitoyens, donneront à l'Union européenne une dimension protectrice et la rendront plus proche des citoyens. C'est dans cet esprit que sera menée la négociation sur la régulation du numérique, qui ne doit pas à elle seule éclipser, ainsi que je le soulignais, l'ampleur du travail accompli sur ce texte. Très bien

du Feader. Ce sont les mesures relatives à la protection des consommateurs sur les plateformes numériques, figurant à l'article 4 , qui ont constitué la pierre d'achoppement. Les députés de la majorité n'ont pas souhaité reprendre ces dispositions,

sur la base du texte que celle-ci avait adopté en octobre dernier en première lecture. Sans surprise, les positions sont restées les mêmes : un accord large sur la plupart des dispositions, mais un désaccord profond et tenace sur l'article 4 , dont la suppression a été maintenue par l'Assemblée nationale. Nous l'avons rétabli en commission la semaine dernière, pour réaffirmer notre point de vue et souligner ainsi ce que nous considérons être une erreur d'appréciation du Gouvernement. Je ne puis imaginer qu'il s'agisse d'une posture de sa part ! Je le dis avec beaucoup de

Je rappellerai tout d'abord que la proposition de loi de Sophie Primas a été adoptée à l'unanimité du Sénat et cosignée par plus de la moitié des sénateurs, sur toutes les travées. L'enjeu est à la fois de conférer davantage de pouvoir au consommateur en ligne, en ouvrant plus largement le champ des possibles, et de donner, par voie de conséquence, plus de place à l'innovation sur des marchés numériques dominés par quelques géants. Le dispositif « clé en main » que nous vous proposons permet de consacrer un principe dit « de de neutralité des terminaux »- c'est très important -et de favoriser l'interopérabilité des plateformes- cela ne l'est pas moins. Il prévoit également de consacrer un article du code de la consommation à la lutte contre les interfaces trompeuses,

? C'est également agir de façon bien différente de ce que vous nous aviez proposé de faire pour la taxation des géants du numérique. J'ajoute que nos amis allemands, eux,

directive transposée. Nous avons donc l'occasion de faire de la France le fer de lance de cette adaptation de notre droit économique à l'économie numérique, en attendant qu'un texte soit adopté au niveau européen dans les années à venir. C'est pourquoi nous nous sommes assez

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme l'iceberg, la majeure partie de l'Union européenne n'est pas dans la lumière. L'Europe fait surtout parler d'elle en période de crise, mais elle ne se résume pas au Brexit. Elle comprend notamment un marché unique, dont bénéficient chaque jour nos concitoyens. Celui-ci est si présent qu'il finit par n'être même plus remarqué. Ce marché commun n'est cependant un progrès véritable que si la concurrence y est loyale, si les règles y sont les mêmes pour tous. Le projet de loi que nous examinons en nouvelle lecture contribue à cette harmonisation, puisqu'il vise à adapter diverses dispositions de notre droit aux règles européennes. En première lecture, le groupe Les Indépendants avait eu l'occasion d'évoquer tout l'intérêt que revêtent les mesures de ce texte, notamment en ce qui concerne les domaines agricole et vétérinaire. Ce texte ne pose d'ailleurs aucune difficulté dans son ensemble. Pourtant, si nous en débattons de nouveau, c'est parce que la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à un accord. La discorde s'est cristallisée sur les dispositions de l'article 4 , c'est-à-dire sur celles qui ont été proposées par la présidente Sophie Primas en vue de protéger le consommateur dans le cyberespace. Je le disais au début de mon propos, l'Union apporte beaucoup aux Européens, mais elle ne fait pas tout. La protection des consommateurs dans le cyberespace reste pour l'instant incomplète. Bien sûr, le, qui sera présenté au début du mois prochain, devrait comporter des dispositions à ce sujet, mais son entrée en vigueur est encore lointaine et pourrait prendre des mois, voire des années.

Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. La France est un acteur essentiel de l'Union européenne. Il est sain qu'elle ne se censure pas dans les initiatives qu'elle peut prendre, au motif que l'Union pourrait s'en saisir plus tard. Notre pays doit assumer sa place et son rôle moteur. Les dispositions proposées par la présidente Primas sont de qualité. Elles ont d'ailleurs été votées à l'unanimité du Sénat, par mon groupe comme par les autres. Le cyberespace est présent depuis plusieurs années dans la vie de nos concitoyens, mais la crise que nous traversons le rend encore plus prégnant. À l'heure où les Français sont appelés à télétravailler le plus possible et où le commerce en ligne devient de plus en plus incontournable, la protection du consommateur en ligne doit être une priorité. Sur internet, le consentement, c'est-à-dire le libre choix du consommateur, n'est pas seulement un enjeu capital des transactions commerciales ; il est aussi un élément majeur de la protection des données personnelles. Nous espérons donc que les dispositions de l'article 4 seront maintenues dans le texte, pour que les Français soient protégés à brève échéance, quitte, le moment venu, à faire évoluer le dispositif au vu des règles européennes. Mon Mon groupe soutiendra l'adoption de ce texte et la protection du libre choix du consommateur dans le cyberespace. La parole

dont les dispositions sont très techniques. De nombreux sujets sont abordés : adaptation de nos règles fiscales et financières, modification de notre droit bancaire, droit des consommateurs, droit commercial, gestion des fonds européens, organisation de notre médecine vétérinaire ... La liste est longue. La France présidera le Conseil européen

mais nous sommes particulièrement gênés par les dégâts que cette façon de traiter une sorte d'inventaire à la Prévert donne à la qualité du débat parlementaire. Pour moi qui entame un premier mandat sénatorial, j'avoue que la découverte d'une telle méthode me laisse perplexe. Si nos gouvernements traitent ainsi, par des listes de courses sans cohérence, le nécessaire travail d'adaptation du droit français aux directives et règlements de l'Union, notre travail et nos débats parlementaires perdront considérablement en consistance et en tenue. Ce texte reflète également la tendance du Gouvernement à privilégier le recours aux ordonnances. Une telle démarche n'est pas de nature à renforcer les liens à nouer entre l'Union européenne et les parlements nationaux, me semble-t-il. à la fin du processus législatif et devons nous prononcer sur l'ensemble de ces articles, qui touchent à des domaines très différents. La commission mixte paritaire a, elle, acté un désaccord. En ce qui nous concerne, nous approuvons les dispositions relatives au secteur vétérinaire, aux droits des consommateurs, au service numérique universel, ou encore aux règles de concurrence et aux télécommunications. Ce texte prévoit des améliorations en matière d'adaptation du droit de la consommation à l'ère du numérique. Il augmentera les capacités d'action de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. Il essaie de faire progresser la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et vise à améliorer l'organisation de la santé animale et du médicament vétérinaire. Nous avons en revanche avec l'article 24 relatif à la gestion du Feader. Cet article prévoit une habilitation à revoir, par ordonnance, la répartition des compétences pour la prochaine programmation pluriannuelle. nous doutons que l'ordonnance soit le meilleur moyen de trouver un accord entre l'État et les régions sur la distribution des fonds européens à nos agriculteurs. Passons du coq à l'âne, puisque ce texte nous y invite. Nous regrettons vivement que l'Assemblée nationale ait supprimé sans autre forme de procès

afin de limiter la croissance externe de ces géants du numérique, qui s'opère par des acquisitions agressives. Enfin, il tendait à protéger les consommateurs contre les interfaces trompeuses. Pour justifier la suppression

Derrière cet acronyme et l'apparente complexité qu'il revêt, ce sont près de dix-huit directives et quatorze règlements européens que nous nous apprêtons à introduire dans le droit français.

le RDSE, par la voix de Josiane Costes, avait insisté sur l'harmonisation des règles financières pour prévenir les infractions relatives au blanchiment, notamment liées au terrorisme. Elle avait aussi mis en avant l'importance du Feader pour nos agriculteurs et nos territoires ruraux. La clarification de la répartition des tâches entre États et régions est la bienvenue. Le transfert vers la région doit être non pas la marque d'un désengagement de l'État, mais celle d'une recherche de subsidiarité, où le niveau le plus efficient- ici la région -doit être compétent, car il est le plus à même de fluidifier l'octroi de ces aides. la première lecture, nous étions parvenus à pointer les réels apports de ce texte concernant la protection des consommateurs sur les plateformes en ligne, que ce soit l'information ou la protection des utilisateurs de réseaux sociaux ou le délai de rétractation face à des pratiques commerciales déloyales. Dans cette période où nos petits commerces sont menacés, c'est adresser un signal important que de sanctionner davantage les fraudeurs et protéger les consommateurs.

concerne l'interopérabilité, mon groupe avait déjà eu l'occasion de souligner son importance lors de l'examen de la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet. Cette faculté d'aller simplement d'une plateforme à l'autre nous permettra, dans un cas comme dans l'autre, de lutter contre les dérives. S'y ajoute un arsenal législatif permettant de lutter contre les interfaces numériques trompeuses, qui, encore aujourd'hui, mettent à mal notre liberté de choix en ligne. Aussi, les arguments de nos collègues de l'Assemblée nationale, qui nous expliquent que l'article 4 serait un cavalier législatif, me convainquent peu. Quel signal envoie-t-on à nos concitoyens lorsque l'on identifie un problème, que l'on trouve une solution pour le résoudre, vote celle-ci à l'unanimité, mais que l'on nous explique qu'elle ne peut être maintenue dans le texte, faute d'examen par l'Assemblée nationale ? Ce qui dérange aujourd'hui nos collègues députés ne les gênait pas il y a deux semaines publique, ou ASAP, dans lequel ce n'était pas un article, mais bien quatre-vingt-un, qui auraient mérité d'être réexaminés de manière classique. Certes, il y a la perspective d'un accord européen, mais personne ne peut dire quand il sera conclu, et la protection de nos concitoyens ne peut plus attendre. Au-delà de ces réserves, il n'y a pas de grands désaccords de fond avec l'Assemblée nationale. Le groupe RDSE, s'il conserve certaines interrogations, votera donc dans sa grande majorité le texte issu de la commission des finances. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'examen des projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne constitue un exercice parlementaire que nous n'apprécions guère trop de sujets essentiels sont réunis dans un même texte, alors qu'ils mériteraient un examen approfondi. Le projet dont nous débattons pour la seconde fois aujourd'hui n'échappe malheureusement pas à la règle. Il touche à de nombreux domaines : droit de la consommation, réglementation financière et douanière, santé animale, transparence dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, droit de la concurrence, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, etc. Sur le fond, certaines Sur le fond, certaines de ses dispositions vont dans le bon sens. Les mesures en faveur de la protection des droits des consommateurs, ainsi que les mesures de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire sont les bienvenues. Celles qui sont destinées à lutter contre les fausses déclarations d'origine douanière des marchandises ou à mieux contrôler les flux d'argent liquide ne peuvent que recueillir notre assentiment.

Vu les délais de transposition- les États membres ont, je le rappelle, jusqu'au 1juillet 2021 pour transposer ces directives, qui seront applicables à compter du 1 janvier 2022 -, il eût été pour nous opportun de soumettre un projet de loi dédié de transposition sur le sujet,

Il n'est pas acceptable de participer à la construction d'une forteresse européenne solidifiée autour des intérêts des marchés financiers et de la spéculation par la libre circulation interne des capitaux. Alors que l'on donne un pouvoir croissant aux acteurs financiers, on a le sentiment d'une « invisibilisation » des États membres dans une union qu'ils subissent trop souvent. Les États doivent pouvoir agir et ne pas avoir les mains liées au nom de principes tels que la concurrence ou la libre circulation des capitaux. Les crises nous montrent l'importance d'une régulation. C'est pourquoi nous ne sommes pas favorables à la transposition, dans ces conditions, des dispositions européennes relatives à la transparence des aides d'État à caractère fiscal. Il ne s'agit pas, comme on pourrait naïvement le croire, de faire en sorte que les citoyens et acteurs économiques soient informés de manière transparente de l'emploi de l'argent public et des allégements de charges accordées aux entreprises ; il s'agit, en réalité, de mieux identifier et contrôler les potentielles atteintes à la libre concurrence et d'éviter que l'État ne soutienne, par des mesures ciblées, un secteur industriel en péril,

l'article 4 propose un nouvel encadrement des géants du numérique, au travers de trois grandes dispositions : la neutralité des terminaux, l'interopérabilité des plateformes et le renforcement du contrôle des concentrations afin d'appréhender les acquisitions dites prédatrices. Après avoir repoussé tout moratoire sur les implantations d'Amazon,

Ce fut le sens du combat mené par le Sénat sur ce texte et, comme l'ensemble de mes collègues, je ne puis que déplorer que le Gouvernement n'ait pas saisi cette chance de proposer une orientation claire,

d'autres avant moi ont expliqué les raisons pour lesquelles nous sommes réunis ici, aujourd'hui, afin de nous prononcer une nouvelle fois sur ce projet de loi. La commission mixte paritaire à laquelle j'ai eu l'honneur de participer s'est réunie le 22 octobre dernier et n'est pas parvenue à un accord.

Cette démarche n'est pas de nature à renforcer les liens indispensables entre les instances européennes et les instances nationales, ainsi que l'articulation de leurs travaux. Cette réserve étant formulée, face à l'urgence de certaines transpositions, nous avions néanmoins accepté l'essentiel des habilitations sollicitées, en précisant parfois leur portée. Sur le fond, ce texte sorti du Sénat et enrichi de nos propositions apparaissait comme globalement positif, au-delà même du fait qu'il permettait la transposition de nombreuses dispositions très attendues. Ces dispositions ayant été déclinées

relatives aux mouvements d'argent liquide en provenance ou à destination des pays tiers et le renforcement des sanctions en cas de violation de la réglementation douanière. Je pense également aux dispositions relatives aux techniques des plateformes numériques de vente en ligne, qui créent des blocages géographiques injustifiés au sein du marché intérieur. Il fallait bien évidemment interdire ces pratiques, pour favoriser la fluidité des marchés dans l'intérêt des consommateurs. Ces dispositions étaient particulièrement souhaitables. Malheureusement, lors de la CMP, nous avons dû faire face à plusieurs points de désaccord, aboutissant, malgré notre bonne volonté, Ainsi, sur l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a rétabli l'article 24 relatif à la répartition future des compétences entre l'État et les régions en matière de gestion du Feader.

Nous n'avons malheureusement pas été écoutés. Mais nous étions prêts à y renoncer, en contrepartie d'une avancée sur les mesures que nous avions introduites dans le projet de loi,

dispositions : la neutralité des terminaux, l'interopérabilité des plateformes et le renforcement du contrôle des concentrations, afin d'appréhender les acquisitions dites « prédatrices » des géants du numérique. Un quatrième dispositif avait été ajouté pour protéger les consommateurs contre les interfaces trompeuses. Ces enjeux sont décisifs, et le Gouvernement avait pourtant indiqué en séance qu'ils étaient au coeur de sa réflexion. Mais il a rejeté l'intégralité des propositions du Sénat, au motif, notamment, qu'elles pourraient créer des distorsions majeures et affecter le dynamisme de l'écosystème des start-up du numérique, pour bon nombre d'entre elles, se développent dans une perspective de rachat par une plateforme plus grande. On ne peut que regretter cette appréciation, d'autant que l'Assemblée nationale a fini par suivre le Gouvernement dans ce rejet de l'article 4 Nous aurions pu ainsi orienter les travaux de la Commission européenne vers une régulation plus agile, plus efficace, qui ne bride ni n'empêche l'innovation et qui permette de mettre un terme à la dynamique actuelle d'enfermement du consommateur. Il semble que l'Allemagne s'engage dès à présent dans cette direction à laquelle nous renonçons

Il est essentiel que la France ouvre la voie en Europe, en attendant qu'une solution européenne soit arrêtée. Oui, c'est au niveau de l'Union européenne qu'il faut agir ! Celle-ci s'est imposée comme un acteur majeur de la régulation numérique, fait preuve de volontarisme sur le dossier. Notre ambition au Sénat est de peser dans les négociations, notamment celles qui auront lieu autour du futur. C'était le sens de nos propositions, qui fixaient un cap et une exigence française.

Aujourd'hui, nous devons faire face à ce rendez-vous manqué, qui aurait été, sans nul doute, un signe encourageant et un soutien à notre gouvernement dans les négociations.

car ils ne concevaient pas une seconde que nos négociations puissent échouer sur un sujet aussi consensuel que la régulation des géants du numérique. Pourtant, au dernier moment, le Gouvernement a tranché : ce sera non ! Non, les consommateurs n'ont pas le droit de recouvrer leur libre choix en matière de smartphone. Non, ils ne pourront pas facilement migrer d'une plateforme à une autre grâce à l'interopérabilité. Non, la lutte contre les interfaces trompeuses n'est pas une priorité. Pourquoi ce non, me direz-vous ? Pourquoi refuser ces nouveaux droits aux Français ? Parce que la Commission européenne a enfin décidé de publier ses propositions sur le sujet en décembre prochain ? C'est la raison avancée par le Gouvernement pour ne pas agir au niveau national. Je souhaite tout d'abord rappeler qu'il n'y a pas de débat entre nous sur la question de savoir s'il faut agir au niveau européen ; très clairement, c'est l'idéal

: il ne faut pas que les parlements nationaux renoncent à leurs prérogatives sous prétexte que la Commission européenne est sur le point de publier une première version Ce serait dangereux, non seulement d'un point de vue démocratique, mais aussi parce que, dans les cas comme celui qui nous occupe, les négociations européennes prennent beaucoup de temps,

Le processus législatif européen est long, et le texte pourrait ne pas être adopté avant plusieurs mois [ ...]. Il est donc indispensable d'agir dans l'intervalle pour responsabiliser davantage les plateformes.

D'un côté, il faut avancer sans attendre l'Europe ; de l'autre, il ne faut surtout pas avancer tant que l'Europe n'a pas entamé son processus législatif.

que l'on entend depuis des années sur le renoncement des élites françaises en matière numérique, sur l'impuissance publique numérique. C'est votre dernière chance. Saisissez-la ! L'histoire et les Français nous regardent,

D'ailleurs, interrogeons-nous : à qui cette situation profitera-t-elle ? Certainement pas aux Français ! Aux quelques firmes américaines concernées, qui, entre nous, n'avaient pas besoin de ce cadeau de la part du gouvernement français.

ce point. Par ailleurs, si la plupart des dispositions étaient issues de textes européens, nous en avons également inséré certaines, par exemple sur les déserts vétérinaires-

La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte de la commission.

pour servir une personne, plutôt que la France

vous pourriez nous dire, monsieur le secrétaire d'État : « Les sénateurs, allez vous coucher, vous n'avez rien compris, la DGCCRF est en train de traiter le problème ! » Mais tel n'est pas le cas. Faites donc ce qu'il faut pour que, dans l'intervalle, entre aujourd'hui et demain,

pas pour vous convaincre- je crois que je n'y réussirai pas -, mais pour enrichir le débat et la connaissance de la Haute Assemblée sur le sujet.

11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. L'article en question traite des cartes de couverture numérique et de prévision de déploiement des réseaux : l'Arcep doit pouvoir demander aux personnes publiques qui exploitent un réseau d'initiative publique ou qui ont élaboré un schéma directeur territorial d'aménagement numérique

les autres dispositions de l'article entrant en vigueur au plus tard le 21 décembre 2023.